Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a souhaité l'inscription de ce débat sur la question, fondamentale des enjeux de la prochaine Parmi les politiques européennes, la PAC tient une place à part. Elle reste en effet, à ce jour, la seule véritable politique européenne intégrée, dotée d'un budget spécifique. Quant à notre pays, il en est aujourd'hui le premier bénéficiaire. Après de premières annonces inquiétantes, l'accord du Conseil européen du 21 juillet 2020 a finalement permis un relatif maintien du budget de la PAC, en euros courants, à hauteur de 386 milliards d'euros. La France bénéficiera ainsi d'une enveloppe stable à hauteur de 62,4 milliards d'euros : 51 milliards sur le premier pilier et 11,4 milliards sur le second. Pourtant, le maintien facial de ce budget cache en réalité une baisse, car, exprimé en euros courants, il ne prend pas en compte l'inflation. Si celle-ci atteint 2 % par an sur la période, on perdrait en réalité 39 milliards, en euros constants, par rapport au budget précédent, soit plus d'une année d'aides du premier pilier. Cette baisse, qui n'est qu'en partie imputable au Brexit, n'est pas un bon signal alors que les défis qui sont devant nous n'ont jamais été aussi grands. Parmi les dix objectifs de cette nouvelle PAC, je retiendrai : assurer un revenu équitable aux agriculteurs agir contre le changement climatique ; garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé ; dynamiser et soutenir le développement économique des zones rurales. Comme vous le voyez, face à de tels enjeux, ce n'est pas le moment de baisser la garde Le plan stratégique national (PSN) est la grande nouveauté de cette future PAC. À partir de 2023, chaque État membre devra obligatoirement mettre en place un PSN qui définira les modalités de mise en oeuvre opérationnelle de la PAC à l'échelle nationale. Nous devrons être très vigilants afin que cette subsidiarité accrue ne fasse pas perdre le sens du « C qui doit être résolument préservé. En effet, si les déclinaisons des PSN revenaient à faire autant de politiques agricoles qu'il y a d'États membres, des distorsions, voire du dumping, pourraient apparaître. Il faut, je le répète, que la PAC reste une politique collective et que tous les agriculteurs, quel que soit leur pays, soient traités sur un pied d'égalité. En outre, le PSN doit garantir que l'agriculture bio ne soit pas la grande oubliée de la future PAC. Actuellement, seulement 2 % du budget de la PAC sont consacrés au bio, ce qui est loin d'être suffisant car, pour atteindre l'objectif de 25 % de terres cultivées en bio en 2030, fixé dans les stratégies Biodiversité et, il faut il faut des mesures fortement incitatives pour transformer les pratiques agricoles. Le PSN, qui conditionnera les règles d'attribution des aides, pourrait donc être le levier pour se rapprocher de l'objectif de 15 % de surfaces en bio en France à l'horizon 2022, que vous aviez réaffirmé, monsieur le ministre, dans le cadre du plan Ambition Bio. Il y en aura besoin car, en 2020, nous en étions seulement à 8,5 %. C'est dans ce sens que nous avons signé une tribune, avec 300 élus locaux et nationaux de différentes sensibilités, sur l'initiative de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique (Fenab), appelant le Gouvernement à intégrer l'objectif du bio dans le PSN. L'autre enjeu de cette nouvelle PAC est une meilleure redistribution des subventions. Le 21 juin 2020, le Conseil a validé le principe d'un plafonnement des aides à hauteur de 100 000 euros par exploitation. Les États membres auront, en outre, la faculté de mettre en place un mécanisme progressif de réduction des aides à partir de 60 000 euros.

Je terminerai par un mot sur les enjeux internationaux de cette nouvelle PAC. Ses objectifs vont dans le bon sens, mais ils sont en complète contradiction avec ce que l'Europe fait, dans le même temps, avec le CETA ( -accord Les normes sanitaires et environnementales que la France et l'Union européenne imposent à nos agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques, faisant de notre agriculture l'une des plus sûres au monde, toujours plus vertueuse en matière de protection de l'environnement. Or ces évolutions ont un coût pour nos agriculteurs en termes d'investissement, de formation et de prise de risque., avec le CETA et le Mercosur, l'Union européenne veut ouvrir le marché européen à des produits alimentaires moins chers, mais qui s'affranchissent des normes sanitaires et environnementales s'imposant à nos paysans. C'est pourquoi je voudrais terminer mon intervention par une question très solennelle, monsieur le ministre : quand aurons-nous enfin un vrai débat avec vous sur ces traités et sur leurs conséquences sur l'agriculture et l'alimentation dans notre pays ? La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis une trentaine d'années, chaque phase de négociation de la PAC constitue une période d'incertitudes pour les professionnels du monde agricole, en particulier pour les éleveurs. C'est précisément la définition des arbitrages pour répartir un budget en baisse qui ouvre le champ à de vives inquiétudes de la part de nombreux territoires et filières. Le 7 avril dernier, vous avez notamment rappelé au Sénat, monsieur le ministre, que la PAC française devait encourager une agriculture de territoires avec une attention portée compensatoire de handicaps naturels (ICHN) et une meilleure prise en compte des zones intermédiaires. Faute, pourtant, d'une définition officielle et unique, l'identification de ces zones intermédiaires, et donc le ciblage de leurs aides, est bien plus difficile que pour les zones défavorisées, qui bénéficient par exemple de l'ICHN. Le critère géographique est lui-même variable selon les appréciations, puisque les pouvoirs publics situent les zones intermédiaires sur une diagonale allant de la Charente au Grand Est. Cette interprétation arbitraire exclut toutefois de nombreux territoires, par exemple dans les régions Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie qui, pourtant, sembleraient être parmi les plus concernées.

Pour atteindre cet objectif, il faudra que la France le finance sur son budget afin de combler la baisse du taux de cofinancement européen de 10 % actée par le Conseil en octobre dernier. C'est un arbitrage qui se défend mais qui aura nécessairement, à enveloppe globale constante, des conséquences sur les autres aides. À cet égard, les zones de polyculture-élevage et les professionnels de l'élevage allaitant craignent que le rééquilibrage de l'enveloppe des aides couplées en faveur de notre autonomie protéique ne se fasse à leurs dépens. Ces aides représentent actuellement 13 % au maximum de l'enveloppe des aides directes, et 2 % pour ce qui est des protéines végétales. Or le Gouvernement envisage une augmentation jusqu'à 4 % des aides dédiées aux protéines afin de renforcer notre indépendance alimentaire et de limiter le recours aux importations. L'objectif est louable, mais les exploitations précitées, qui ont déjà été, pour certaines, sorties du dispositif de l'ICHN et demeurent fragiles, ne pourront pas supporter de nouvelle diminution. Par exploitation, le montant des aides allouées correspond à peu près au salaire mensuel des éleveurs, c'est-à-dire 800 euros par mois. Si rééquilibrage il doit y avoir, celui-ci devra engager financièrement les filières agricoles les moins impactées par la crise. Par ailleurs, notre groupe attend des avancées sur le sujet des paiements redistributifs et sur la convergence des aides. Si rien n'est encore acté, je tiens tout de même à rappeler que ces aides couplées bénéficient pour 80 % à l'élevage. La Fédération nationale bovine (FNB) s'est fait l'écho de cette préoccupation, en demandant que les aides couplées du premier pilier soient impérativement maintenues à leur niveau actuel. Il y va de la survie de nombreuses exploitations et donc, plus largement, de l'équilibre économique mais aussi environnemental de nombreux territoires ruraux. L'élevage extensif qui les caractérise contribue, grâce aux prairies permanentes, à la captation du carbone et permet l'approvisionnement des agglomérations proches des exploitations en produits de qualité des circuits courts.

un soutien massif en faveur de ce modèle agricole. D'autre part, une question demeure concernant l'augmentation de notre autonomie protéique : visera-t-elle en priorité l'alimentation animale ou humaine ? Sur ce point, les éleveurs manquent de précisions, surtout au regard du souhait du Gouvernement de pérenniser les repas végétariens hebdomadaires dans les cantines scolaires. Face à ces multiples impératifs- préserver notre modèle d'élevage extensif et augmenter notre autonomie protéique -où placer le curseur ? Comment arbitrer ? Monsieur le ministre, il faut selon moi, avant tout, déterminer quel modèle agricole et Un modèle qui promeut des pratiques, tant d'élevage que de culture, vertueuses et respectueuses de l'environnement, des animaux et des hommes ? Ou un modèle d'agriculture intensive dont on ne cesse de rappeler les multiples effets dévastateurs ? Une fois ce choix fait, les arbitrages devraient logiquement en découler. en découler. Pour une fois, faites en sorte que les éleveurs ne soient pas les seuls à porter l'effort budgétaire, alors que leur situation ne le permet pas. Pouvez-vous nous assurer que les zones de polyculture-élevage ne seront pas les sacrifiées de la future PAC ?

après la gelée noire subie dans la nuit du 8 au 9 avril par un grand nombre d'exploitations en France et compte tenu de mes travaux depuis 2016 sur ce sujet, je n'aborderai qu'un seul thème : celui de l'assurance récolte. La gestion des risques- nous en sommes désormais tous convaincus -est centrale pour l'avenir de notre agriculture. En France, les filières se sont engagées dans des modes de production durables. L'Europe, la future PAC, a conditionné les aides à des objectifs de verdissement. Ces mutations répondent à la demande sociétale et aux enjeux de santé publique et de protection de l'environnement. Mais encore faut-il accompagner notre agriculture dans sa résilience. Celle-ci doit s'appuyer sur plusieurs solutions : l'épargne de précaution, les mesures de stockage, les outils de stabilisation des revenus et l'assurance récolte.

Or la PAC demeure un levier d'accompagnement majeur de l'agriculture. Je conçois que l'exercice soit complexe, et que les aides du premier pilier soit structurantes pour l'économie d'un grand nombre d'exploitations agricoles. Permettez-moi un maraîcher qui exploite un hectare et emploie cinq salariés perçoit 5 000 euros de PAC quand un céréalier qui exploite 5 000 hectares percevra 1 million

de subsidiarité et la possibilité pour la France de moduler et de plafonner elle-même ses aides.

à mon sens, pourrait être mieux définie et relever de la compétence et des choix politiques de l'État français.

Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé publiquement à plusieurs reprises en faveur du maintien en l'état de l'enveloppe consacrée à l'ICHN dans la nouvelle PAC. Malgré cela, le taux de cofinancement européen proposé par le Conseil passe de 75 % à 65 %. Si ce taux était définitivement retenu et si la France décidait de maintenir l'enveloppe actuelle, elle devrait financer sur son budget 10 % supplémentaires, soit environ 108 millions d'euros. Dans le contexte de la négociation qui va s'ouvrir demain à enveloppe fermée, quels arbitrages comptez-vous faire pour financer ces 108 millions d'euros, si bien entendu vous comptez le faire ? second volet est lié aux conséquences de la sortie du zonage des zones défavorisées dites « simples ». Ce zonage a fait l'objet d'une révision en 2018. Celle-ci a eu pour effet d'exclure 1 350 communes de la cartographie, laquelle fut présenté à la Commission européenne

éviter l'effet ciseaux. Qu'en est-il ? Dans l'Aude, rien, nada : l'ICHN a bel et bien disparu, mais aucune des promesses faites n'a été tenue. Quel dispositif avez-vous prévu pour aider, soutenir ces agriculteurs et ces éleveurs qui ne demandent qu'à vivre dignement de leurs exploitations ? monsieur le ministre.

au sein du Conseil et du Parlement européens. Le Sénat a effectué pour sa part un important travail de réflexion et de proposition. Ainsi, trois propositions de résolution européenne ont été adoptées en 2017, 2018 et 2019, les deux dernières en séance publique et à l'unanimité. Au-delà de la question de la stabilité des moyens budgétaires, nous nous sommes vivement inquiétés de l'architecture générale du projet de la Commission européenne, notamment de l'impact du nouveau mode décentralisé de mise en oeuvre de la PAC. Décentraliser la PAC, c'est prendre le risque de distorsions de concurrence supplémentaires au sein du marché unique. Le Sénat y voit un réel danger de remplacement de la PAC par vingt-sept politiques agricoles nationales, désormais de moins en moins compatibles entre elles. En dernière analyse, nous courons le risque d'une déconstruction de la PAC. Or, sur tous ces points essentiels, la position de la Commission européenne n'a pour ainsi dire jamais changé d'un iota. Depuis 2017, vos prédécesseurs, monsieur le ministre, n'ont pas agi à temps et efficacement pour faire bouger les lignes. Cette réforme ne correspondra donc guère aux voeux du Sénat ni aux besoins de nos agriculteurs dont l'inquiétude va croissant. Reste désormais à clarifier un problème de fond : celui de l'articulation entre les modalités détaillées de la future PAC et la transcription juridique des objectifs affichés dans la transition verte.

Comment, selon vous, articuler la réforme de la PAC et le si l'on veut éviter un recul drastique de la production agricole européenne à l'horizon 2030, recul que le ministère américain de l'agriculture évalue pour sa part à 12 % ? à 12 % ? Autre question de taille : face à une perspective de décroissance d'une telle ampleur de nos productions nationales, que deviendrait l'objectif de souveraineté alimentaire ?

le changement climatique, la pandémie de covid-19, les défis de souveraineté et d'alimentation ... L'agriculture est, depuis toujours, synonyme d'adaptation. Je voudrais faire remonter les craintes de nos agriculteurs de zones très rurales au sujet de la future PAC.

Il en ira très vraisemblablement de même de l'objectif d'intégration de 20 % de produits bio dans la restauration collective, voté dans la loi Égalim. Des importations ! Pourtant, malgré ces échecs, le Gouvernement continue de baisser l'accompagnement financier à cette agriculture. Après la fin du financement national de l'aide au maintien, c'est aujourd'hui la réforme de la PAC qui acte un nouveau recul. Alors que la performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture biologique est établie, alors que la demande des consommateurs ne cesse de croître, ne cesse de croître, alors que l'urgence écologique est toujours plus prégnante, les premières propositions du PSN montrent que la bio sera la grande perdante de cette réforme. D'après les chiffres qui sont sur la table des négociations,

comment expliquez-vous une telle diminution du soutien au maintien en agriculture biologique, alors même que la rémunération des services environnementaux faisait partie des engagements présidentiels ?

proposer un scénario alternatif permettant d'atteindre les objectifs de la France et de rémunérer ce système à la hauteur de ses performances économiques et écologiques

mais beaucoup d'agriculteurs restent aussi oubliés de la PAC. Je pense aux petites fermes, aux maraîchers, aux arboriculteurs, aux paysans herboristes, qui sont en marge du système et qui ne sont pas pris en considération, alors qu'ils assurent la résilience, l'emploi et le respect de l'environnement. La parole

l'agriculture est un secteur stratégique, qui se situe aujourd'hui au carrefour de nombreux enjeux. En plus de devoir assurer notre souveraineté alimentaire, il doit répondre à une exigence croissante de qualité. Il s'agit aussi pour la profession de s'orienter vers une agriculture plus durable, respectueuse de l'environnement et soucieuse du climat. Répondre à ces enjeux nécessite de la part des agriculteurs qu'ils réalisent de gros efforts, alors même qu'ils sont déjà soumis à de nombreuses contraintes telles que la multiplication des aléas climatiques ou encore la volatilité des prix. Dans ce contexte, les négociations en cours concernant la PAC constituent un enjeu de taille pour notre pays et ses agriculteurs. À ce titre, nous savons tous que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour placer la France au coeur des enjeux européens, ce qui a permis à la PAC de demeurer le premier budget européen, et à notre pays de conserver l'enveloppe qui lui était allouée. Ces aides de la PAC, sans lesquelles beaucoup d'agriculteurs auraient des revenus négatifs, doivent les encourager sur le chemin de ces mutations. Les contours encore flous de cette nouvelle PAC suscitent toutefois des inquiétudes chez les agriculteurs. Ils craignent notamment qu'une mise en oeuvre différenciée des objectifs de la politique européenne au travers des PSN n'aboutisse à des situations de distorsion de concurrence entre États membres. Ils se soucient également des critères d'accès aux écorégimes, qui doivent être aussi inclusifs et incitatifs que possible. Comment entendez-vous répondre à ces inquiétudes ? Plus largement, comment préserver la compétitivité et la rentabilité de notre agriculture tout en encourageant sa mutation vers un modèle plus durable et plus raisonné ?

monsieur le ministre. Venant d'un territoire frontalier, l'Alsace, je tenais encore à insister sur les inquiétudes en termes de concurrence que pourraient engendrer les mesures de la future PAC. Le risque de concurrence déloyale existe à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, mais aussi à ses portes. Aussi, nous comptons sur vous, avec l'Europe, pour veiller à ce que les importations extraeuropéennes répondent à des exigences qui soient au moins équivalentes à celles que nous imposons à nos agriculteurs. Il y va de la survie de notre agriculture.

elle produit souvent des produits de qualité. Pourtant, lundi dernier, au marché de Valence-d'Albigeois, les veaux se sont vendus au même prix qu'il y a trente

monsieur le ministre,

que le soutien à une agriculture de territoire de montagne avec une meilleure prise en compte des spécificités et le maintien de l'ICHN était l'une des priorités de la nouvelle PAC. Élu d'un territoire de montagne, je ne peux que souscrire à cette volonté, qui permet de maintenir un maillage d'actifs agricoles et une présence humaine dans ces territoires. C'est le plus sûr moyen d'empêcher l'abandon des terres et leurs conséquences négatives en termes de paysage, de biodiversité et de développement, notamment touristique. La PAC 2023-2029 introduira une innovation en termes de gouvernance, à travers les PSN, qui renvoient à chaque État membre le soin de définir les modalités de mise en oeuvre de la PAC à l'échelle nationale. Vous aurez donc, monsieur le ministre, à décider du soutien que vous accorderez à l'agriculture de montagne.

pour compenser la baisse européenne annoncée ? J'ai entendu que vous vous engagiez à hauteur de 140 millions d'euros par an. J'espère que cette promesse sera tenue Pouvez-vous aussi nous confirmer que les surcoûts des exploitations de montagne liés aux handicaps naturels continueront d'être compensés au moins à leur niveau actuel, au travers d'une ICHN forte qui ne subira pas de baisse ? ? Et qu'en est-il de possibles extensions à certaines productions végétales ? Enfin, monsieur le ministre, si nous appelons de nos voeux une meilleure gestion et prise en charge des risques climatiques, il ne faudrait pas non plus que de nouvelles mesures viennent diminuer les aides existantes.

Pourtant, chacun s'accorde à dire combien elle est nécessaire pour répondre aux enjeux complémentaires et parfois contradictoires qui permettent d'assurer notre sécurité alimentaire, tout en renforçant les actions favorables à l'environnement mais aussi au tissu socioéconomique des zones rurales. À cet égard, une évidence se fait jour : la France doit effectuer des propositions qui vont dans le sens de la simplification, en rendant la PAC plus accessible et plus lisible. Dans cette perspective, elle se doit de construire l'architecture des PSN autour de celui qui fait l'agriculture : l'agriculteur.

avec des approches et des pratiques différentes. Il se doit d'être accompagné dans la réalité de son métier pour percevoir une juste rémunération. Il en va de la reconnaissance de la valeur travail comme du nécessaire renouvellement des générations. Au regard de l'évolution du métier, du revenu, de la main-d'oeuvre occupée sur l'exploitation et de l'objet social, au regard de ceux qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, au regard des spécificités des surfaces et des territoires- je pense là aux zones de châtaigneraies, de chênaies, ou encore aux zones humides de Camargue, dans le département du Gard, qui sont encore soumises à dérogation -, pourrions-nous définir, afin de le protéger, un statut de l'agriculteur ? Pouvons-nous compter sur vous, monsieur le ministre, pour porter l'exigence de cette clarification et intégrer cette question dans les prochaines échéances ? La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crises sanitaires et les dérèglements climatiques mettent en évidence la nécessité de repenser nos modèles économiques et de développement. Construire des circuits courts, économes en énergie, de la production à l'assiette à l'assiette du consommateur, élaborer des process de qualité, entretenir et améliorer chaque jour le cadre naturel et environnemental, tels sont aujourd'hui les principaux axes de travail pour tous les États membres de l'Union européenne, à l'heure où nous discutons de la Le modèle d'exploitation agricole français s'est construit à partir d'unités de production de taille modeste, souvent familiales et transmises sur plusieurs générations. Alors que beaucoup jugeaient ce modèle

Monsieur le ministre, je sais que les équilibres sont complexes et que les exploitations agricoles ont des tailles diverses. Pour autant, nous avons absolument besoin d'une PAC sociale, pour soutenir les femmes et les hommes

Alors que les agriculteurs ont un genou à terre, nous devons les aider à se relever », écriviez-vous. La question que je souhaite vous poser ce soir est celle que se posent en fait les éleveurs de viande charolaise de mon département de la Saône-et-Loire

Trois ans après la loi Égalim, les éleveurs de bovins ont perdu 30 % de leurs revenus, pour se contenter désormais de moins de 700 euros par mois en moyenne, ces maigres revenus correspondant justement aux aides de la PAC qui leur sont versées ... Diminuer ces aides signifierait réduire encore leurs revenus.

bétail, l'UGB, que vous souhaitez instaurer sera-t-elle la même pour les bovins laitiers et les bovins allaitants ? Quel en sera le montant ? Allez-vous les plafonner à 100 UGB ? En effet, les plafonner, ce serait condamner plusieurs milliers d'exploitations de Bourgogne-Franche-Comté à une chute des aides En cas de baisse importante de ces aides, comment éviterez-vous une décapitalisation violente dans les élevages, avec les conséquences que l'on imagine sur les prix et la filière ? Ce ne sont pas là, monsieur le ministre, des « carabistouilles », pour reprendre votre expression, mais des questions empreintes d'inquiétude, qui appellent des réponses précises et chiffrées. La parole est à M.

la filière betteravière est aujourd'hui en réel danger. Vous insistez régulièrement sur la question de la souveraineté alimentaire de notre pays ; cette filière y participe, et les enjeux sont aussi agricoles qu'industriels. Il faut répondre à cette urgence, et il est essentiel que le plan stratégique national de la PAC comporte un volet de nature à sécuriser, conforter et relancer la filière de la betterave. Au-delà de la question des dispositifs des premier et deuxième piliers et de l'accompagnement de la structuration des filières, les professionnels en appellent à une stratégie sectorielle de gestion des risques, complémentaire du développement de l'assurance récolte. Ils soutiennent également la mise en oeuvre d'un instrument de stabilisation qui serait de nature à conforter les revenus des betteraviers face au choc économique et aux sinistres sanitaires non éligibles au Fonds national Monsieur le ministre, que prévoit le Gouvernement, en termes de priorités, de dispositifs et de moyens, dans le cadre de la prochaine PAC, pour sauvegarder et relancer la filière betteravière ?

Monsieur le ministre, les objectifs de la PAC 2021-2027 sont posés : favoriser une agriculture assurant souveraineté et santé alimentaire ; développer les actions favorables aux objectifs environnementaux et climatiques fixés par l'Union européenne ; renforcer le tissu économique des zones rurales. Depuis 2014, la convergence progressive des aides a eu pour conséquence une forte baisse des aides directes pour certaines régions, dont les Hauts-de-France, au profit d'autres régions. La moyenne par exploitation dans la Somme, par exemple, a diminué de 42 % en dix ans. En 2014, le paiement redistributif, passé de 5 % à 10 %, a permis à certaines régions de compenser pour partie cette convergence du paiement de base. Tel ne fut pas le cas dans la Somme, qui, de plus, comme d'autres départements, ne bénéficie pas des indemnités compensatoires de handicaps naturels, les ICHN, du second pilier. Les importants transferts du premier pilier au second pilier ont donc eu un impact négatif sur les paiements de base dans ces territoires. La convergence progressive aujourd'hui proposée à 80 % correspond, dans la Somme, à une nouvelle diminution de 12 euros par hectare, soit 5,66 millions d'euros. Et, si la convergence était de 100 %, elle serait de 8,5 millions d'euros. d'euros. Dans le cadre du plan stratégique national, le PSN, vous devez, entre autres objectifs, définir les quatre modalités de la convergence interne du montant de paiement de base : convergence nationale ou régionale ; seuil de déclenchement de la convergence ; écart à la moyenne comblée par convergence ; limitation ou non et compensation ou non des pertes suscitées par la convergence. Monsieur le ministre, quelles garanties apportez-vous sur le montant du premier pilier et sur le transfert ou non des montants du premier au second pilier permis par le règlement ? Quelle convergence, quel taux et quel calendrier envisagez-vous ? Par ailleurs, pour limiter la compensation des pertes successives pour les systèmes de production des grandes cultures, dont dépendent les filières industrielles, comme le blé, le protéagineux ou la betterave, permettrez-vous un accès aux écorégimes simples à tous les modèles de production, avec la prise en compte des évolutions agroéconomiques, comme la gestion de l'eau ou l'agriculture de précision, et quelle convergence des droits sera appliquée Enfin, dans le cadre de la convergence, à quel niveau allez-vous fixer la part du paiement redistributif, dont on sait qu'il est, certes, un facteur de convergence des aides découplées, mais dont le doublement de la part, de 10 % à 20 % du montant du premier pilier, entraînerait, dans la Somme, une perte supplémentaire de 5 euros à 10 euros l'hectare

Cette inquiétude est très légitime au regard des nombreux points de désaccord et de la très lente progression des négociations en trilogue sur la réforme de la PAC. Et elle est renforcée dès lors que l'on mesure les conséquences que pourraient avoir des arbitrages sur les équilibres fragiles de certaines exploitations. En Haute-Saône, monsieur le ministre, plus de 80 % de la surface agricole utile est en zone défavorisée, caractérisée par des sols superficiels, voire très superficiels. Pour pallier ces handicaps, les efforts sont incontestables. En polyculture-élevage, les agriculteurs développent des systèmes particulièrement autonomes, résilients et vertueux sur le plan environnemental, qui méritent une attention toute particulière. La politique agricole commune, au travers du second pilier, soutient et accompagne ces exploitations situées en zone défavorisée. Or la PAC va changer, mais les contraintes de production, elles, ne changent pas ; elles ont même Si la faible qualité des sols est presque routinière pour nos paysans, le fléau de l'excès de sécheresse est une calamité à laquelle on ne se fait pas. Dans ce contexte, un changement brutal de paradigme serait un coup mortel porté à nos agriculteurs, dont les revenus sont au plus bas, et, en cascade, à nos paysages et à notre biodiversité. Pour éviter ce désastre, une prise en considération totale de l'ICHN s'impose en faveur des zones défavorisées simples, en Haute-Saône notamment. Il importe aussi de reconnaître certaines spécificités, comme celles des zones intermédiaires. L'État devra également s'engager à compenser la baisse des cofinancements du Fonds Monsieur le ministre, dans quelle mesure ces spécificités territoriales seront-elles prises en compte ? En d'autres termes, quelle « agriculture des territoires » attend demain ces paysans des terres à handicap

j'aurai la certitude d'avoir fait ces choix avec le plus de concertation et de professionnalisme possible. C'est un engagement de moyens et pas forcément de résultats. Pardonnez-moi de me contredire par rapport à ma réponse de tout à l'heure, monsieur le sénateur, mais je crois que c'est ainsi que l'on fait avancer les choses, en tout cas dans le cadre d'un PSN, avec, et je veux les remercier, des services qui, derrière moi, travaillent jour et nuit depuis de nombreux mois sur cette question pour mener ces concertations, qui ne manquent

Dans ce moment inédit de mise au point du plan stratégique national, le PSN, dont l'issue aura de lourdes conséquences pour nos agriculteurs et nos territoires, et en m'inspirant des mots du philosophe- « Que puis-je connaître ? Que m'est-il permis d'espérer ? Que dois-je faire ? » je vais m'attacher à conclure ce débat. Tout d'abord, nous connaissons le budget dont bénéficiera la ferme France. Le contexte du cadre financier pluriannuel était difficile avec le départ des contributeurs nets. Il est facialement équivalent à celui de la période précédente, mais il sera en baisse en euros constants, seule unité de mesure sérieusement utilisable pour comparer des budgets sur longue période.

les agriculteurs français doivent tous pouvoir vivre décemment de leur métier. La Nation doit leur assurer un revenu équitable, tout en répondant aux attentes de la société en matière de qualité, de santé et d'impact sur l'environnement et le climat. Avec un budget en baisse et des marchés que nous ne maîtrisons pas- il s'agit d'un sujet que nous n'avons pas abordé -, où va-t-on trouver les moyens de répondre à cet objectif ? Tout d'abord, il faut rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Égalim première version a été, malgré nos avertissements de l'époque, un échec. Il est urgent de rouvrir le débat sur la base d'une construction du prix payé par le premier acheteur, intégrant des critères de coûts de production dans un cadre contractuel pluriannuel. tout l'inverse du ruissellement, dont le premier des Américains vient de nous dire qu'il n'a jamais marché ... Les paysans français l'avaient compris depuis longtemps à leurs dépens. Il aurait certainement fallu les écouter ! Et que dire aux agriculteurs qui ont été injustement et dramatiquement sortis de la carte des zones défavorisées ?

Ne faites pas l'erreur de jouer les protéines contre l'élevage allaitant. La réforme de l'unité de gros bétail, l'UGB, doit apporter aux éleveurs, et non pas les affaiblir À enveloppe constante, nous pensons qu'il faut cibler les aides sur les systèmes productifs à enjeu, comme le bio, l'agriculture de conservations des sols, les démarches de qualité certifiée, RSEA, sans oublier les appellations et autres marques de pays. Garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé en réponse aux attentes de la société passe indéniablement par ces démarches, qu'il faut soutenir davantage.

à travers la mise en place de paiements pour services environnementaux, ou PSE. Plus largement, la notion d'aménités rurales doit se traduire par une meilleure reconnaissance de la place de la ruralité dans notre pays. C'est un enjeu national, qui déborde le strict cadre de l'agriculture. Monsieur le ministre, nous vous demandons

Il y va aussi de la dynamisation et du soutien au développement des zones rurales. Les collectivités locales y auront toute leur place, en lien avec l'agenda rural. La question cruciale du renouvellement des générations passera par là. La définition de l'actif agricole et des nouvelles dispositions de gestion du foncier agricole y contribuera également grandement. Nous souhaitons en outre que votre feuille de route sur les zones intermédiaires, les ZI, puisse prendre en compte la diversité des territoires en difficulté. Les ZI ne se limitent pas à la diagonale « Charente-Maritime-Moselle

Le revenu et la compétitivité passeront aussi par la protection et la création de ressources naturelles, au premier rang desquelles nous plaçons la ressource en eau. Vous avez ouvert le dossier, et nous sommes disponibles pour travailler avec vous sur ce sujet majeur et urgent, qui ne concerne pas que le sud de la France. Il faudra donc améliorer la compétitivité sans sacrifier les enjeux de qualité alimentaire, de santé et d'impact des productions sur l'environnement.

Pour conclure, je dirai un mot sur les enjeux internationaux de la PAC pour notre pays. Monsieur le ministre, nous vous demandons de faire en sorte que les producteurs français soient traités équitablement, donc que les critères d'exportation soient équivalents aux critères d'importation et intègrent notamment la problématique du carbone et des normes sanitaires. Je vous